J'informe le Sénat qu'une candidature pour siéger au sein de la commission des affaires européennes a été publiée. Cette candidature sera ratifiée si la présidence n'a pas reçu d'opposition dans le délai d'une heure prévu par notre règlement. Mes chers collègues, en raison de l'hommage national en l'honneur de Samuel Paty, qui se tiendra mercredi 21 octobre en fin d'après-midi dans la cour de la Sorbonne, en accord avec le groupe du Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, nous suspendrions nos travaux demain après-midi à l'issue de l'examen de la proposition de loi relative à la déshérence des contrats de retraite supplémentaire, les reprendrions à vingt et une heures trente pour le débat à la suite du Conseil européen des 15 et 16 octobre. Il reviendra à la conférence des présidents d'inscrire le débat sur l'alimentation durable et locale, initialement inscrit en second point de l'espace réservé au groupe du Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants,

Par ailleurs, par lettre en date de ce jour, le Gouvernement demande l'inscription, sous réserve de son dépôt et de sa transmission, du projet de loi autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses dispositions de gestion de la crise sanitaire à l'ordre du jour du mercredi 28 octobre,

En conséquence, l'examen du projet de loi de programmation pluriannuelle de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur est reporté aux jeudi 29, l'après-midi et le soir, et vendredi 30 octobre, le matin, l'après-midi et, éventuellement, le soir. Acte est donné de ces demandes. Nous pourrions fixer le délai limite pour le dépôt des amendements de séance en première lecture sur le projet de loi autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire au mercredi 28 octobre à En cas de nouvelle lecture, le délai limite pour le dépôt des amendements de séance pourrait être fixé au jeudi 5 novembre à douze heures. Y a-t-il des observations ? ... Il en est ainsi décidé. Mes chers collègues, pour le respect des règles sanitaires, je vous rappelle que le port du masque est obligatoire dans l'ensemble du palais. Il vous est demandé de laisser un siège vide entre deux sièges occupés. L'hémicycle fait l'objet d'un nettoyage et d'une désinfection chaque semaine ; les micros sont régulièrement désinfectés. J'invite chacune et chacun d'entre vous à veiller au respect des distances de sécurité. Je rappelle également que les sorties de la salle des séances devront exclusivement s'effectuer par les portes situées au pourtour de l'hémicycle. Enfin, afin de limiter la circulation de documents, vous êtes invités à utiliser vos tablettes et la fonctionnalité « En séance » sur le site internet du Sénat pour prendre connaissance du dérouleur et des amendements. L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi constitutionnelle et de la proposition de loi organique pour le plein exercice des libertés locales, présentées par MM. Philippe Bas et Jean-Marie Bockel et plusieurs de leurs collègues

de décentralisation, qui leur incombait au sein de la commission des lois. Au début de cette année, le président du Sénat, Gérard Larcher, a réuni un groupe de travail. J'en étais le rapporteur général ; Jean-Marie Bockel, que je salue- il a quitté le Sénat, mais son travail mérite d'être reconnu -, en était le corapporteur. Nous avons abouti à un document publié par le président du Sénat

Madame la ministre, vous vous demandez peut-être pourquoi nous avons voulu commencer- ce n'est pas le cas de votre projet de réforme -par une réforme d'ordre constitutionnel. Je me permets de le souligner

Ce fut le cas en 2003, lors de l'étape franchie sur l'initiative du président Jacques Chirac et de son Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin, pour le renforcement de la décentralisation. Ce devrait être le cas aujourd'hui, à condition que le Gouvernement soit, comme nous, animé d'une ambition forte pour les libertés locales

deuxième point, c'est d'empêcher que l'État ne récupère les pouvoirs qu'il décentralise. C'est la pratique française

n'a cessé d'agir pour récupérer les pouvoirs qui étaient décentralisés. Comment a-t-on procédé en France ? Très simplement : par la norme et par l'argent. Les normes se sont multipliées ; l'autonomie financière des collectivités locales n'a cessé d'être rognée, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Le troisième point, c'est de garantir l'indépendance financière des collectivités

Le quatrième point, c'est de permettre à chaque catégorie de collectivités territoriales d'avoir des compétences à géométrie variable, autour d'un tronc commun. Il faut mettre un terme à cette uniformité bien française qui stérilise les initiatives.

Pour construire l'avenir sur des fondations solides, nous proposons plusieurs éléments d'ordre constitutionnel. nous voulons renforcer le pouvoir réglementaire des collectivités territoriales. Selon nous, l'intervention du décret dans la mise en oeuvre des compétences que le législateur donne aux collectivités territoriales devrait être l'exception. La règle devrait être l'exercice, par les collectivités, de leur pouvoir réglementaire,

le cas. De surcroît, il me paraît extrêmement important de garantir une représentation équitable des territoires dans les assemblées locales, en particulier les intercommunalités.

les attentes exprimées par les représentants de chaque territoire. Quand, au sein d'une intercommunalité, on s'entend pour répartir

Nous voulons aussi consacrer dans la Constitution la clause générale de compétence des communes. Je le disais : prenons garde à ce que la commune ne devienne pas une coquille vidée dans l'intercommunalité. Il est très important que les communes se considèrent comme les actionnaires de l'intercommunalité, et non pas comme ses sujets. Pour ce faire, Pour ce faire, il nous paraît essentiel de préserver leur clause de compétence générale, quelle que soit la manière dont elles choisissent de l'exercer : elles peuvent bien sûr choisir de déléguer la compétence au niveau intercommunal. Madame la ministre, nous voulons également instituer un droit à la différenciation.

dans un cadre juridique beaucoup plus souple que le cadre constitutionnel actuel. Mes chers collègues, cet ensemble de dispositions constitutionnelles est extrêmement important. Il est sans doute plus important encore que les deux précédentes révisions constitutionnelles, que j'ai citées, en matière de décentralisation. Ces dispositions sont complétées par plusieurs propositions relevant de la loi organique. Ces dernières visent, d'une part, à circonscrire le périmètre des ressources propres aux impositions de toutes natures dont les collectivités territoriales fixent l'assiette, le taux ou le tarif et, d'autre part, à renforcer les études d'impact. Cette exigence constitutionnelle fondamentale a été vidée de sa substance

et la proclamation solennelle, dans la Constitution, de l'organisation décentralisée de la République. Le second a été un temps en arrière, avec la reprise en main des collectivités par l'accumulation des normes et la mise sous dépendance des finances locales.

avec les dispositions spécifiques aux territoires d'outre-mer et, plus récemment, avec la création de la collectivité européenne d'Alsace, ou encore, dans ma chère Bretagne, avec la territorialisation du dispositif d'investissement locatif pour le logement. Niez le réel, et il vous revient au visage comme un boomerang ! La crise sociale des « gilets jaunes » a révélé un besoin criant de proximité et de confiance. La crise sanitaire a prouvé et prouve encore le sens des responsabilités, la réactivité et l'agilité des collectivités locales. Elle a également montré l'impuissance d'une gestion de crise centralisée, avec un État ankylosé par de trop grandes rigidités. Le Sénat, représentant des collectivités territoriales, ne cesse d'affirmer que l'action publique ne peut trouver son efficacité qu'en inversant notre logiciel : il faut construire à partir du principe de subsidiarité, décider de faire au niveau pertinent. C'est dans cet esprit que le président du Sénat a constitué, au premier semestre, un groupe de travail réunissant tous les groupes politiques. Je salue le travail accompli par les deux corapporteurs, M. Philippe Bas, alors président de la commission des lois,

et à consacrer la pleine reconnaissance des responsabilités locales. Nous examinons aujourd'hui les volets constitutionnel et organique de ces textes, qui visent à permettre un rééquilibrage des pouvoirs entre l'État et les collectivités locales sans toutefois provoquer un nouveau « big-bang territorial Il s'agit de permettre et non plus de contraindre. Avant de céder la parole à Mathieu Darnaud, je tiens à exposer quelques-uns des objectifs retenus. Le premier objectif est de consacrer dans la Constitution la représentativité équitable des territoires. par deux apports : inscrire le terme « territoire » dans la Constitution et redéfinir la représentation proportionnelle pour les collectivités locales,

est d'adapter les compétences des collectivités à leurs réalités locales en renforçant le pouvoir réglementaire local et en inscrivant dans la Constitution le droit à la différenciation. la possibilité de pérenniser les expérimentations locales sur une partie seulement du territoire et la possibilité, pour le législateur, d'attribuer des compétences distinctes à des collectivités territoriales de même catégorie. de loi organique, elle vise, par son article 1, à renforcer les études d'impact- je sais que certains de nos collègues sont très sensibles à cet enjeu -afin que le législateur puisse légiférer plus sûrement et en parfaite connaissance de cause. de loi visent à sécuriser les compensations financières des transferts de compétences de l'État aux collectivités, selon le principe « qui décide paie ». Nous pensons tous, et ce n'est qu'un exemple, aux difficultés engendrées, pour les départements, par le

Toute crise offre des occasions à saisir. Tirons ensemble les leçons de la mobilisation des collectivités territoriales, fortes et responsables. N'ayons pas peur. Osons emprunter le chemin de la confiance et des libertés locales : c'est celui de la réussite, pour sortir notre pays de ses lourdes difficultés ! La parole

comme le premier des échelons administratifs, mais plus encore comme un lieu où se tisse le lien social, comme le creuset de toutes les solidarités. La crise sanitaire que nous vivons nous rappelle, jour après jour, la nécessité de défendre la commune.

nous examinons aujourd'hui deux propositions de loi, l'une constitutionnelle, l'autre organique, pour le plein exercice des libertés locales. Ces textes ont été déposés, notamment, par nos collègues Philippe Bas et Jean-Marie Bockel et font suite aux conclusions du groupe de travail sur l'avenir de la décentralisation, présidé par Gérard Larcher. Parmi l'ensemble des mesures que comportent ces propositions de loi, deux ont justifié que la commission des finances se saisisse : c'est sur ces dispositions que je m'exprimerai. La première est la révision des modalités de compensation des charges transférées aux collectivités territoriales, avec la consécration du principe « qui décide paie ». La seconde est la redéfinition du périmètre des ressources propres des collectivités territoriales.

Mais, comme la commission des lois, j'ai estimé que le dispositif de réévaluation proposé pouvait être amélioré. À mon sens, ce qu'il faut chercher à construire, c'est une gouvernance nouvelle par laquelle l'adéquation des ressources et des charges des collectivités territoriales serait régulièrement réinterrogée.

c'est une bonne chose de construire un espace de dialogue entre l'État et les collectivités locales. Celui-ci permettra de remettre à plat régulièrement les compétences et les compensations.

des simulations ont été effectuées pour estimer l'impact qu'aurait la mise en oeuvre d'une redéfinition des ressources propres excluant les recettes fiscales sur lesquelles les collectivités territoriales n'exercent aucun pouvoir de taux ou d'assiette. Il va sans dire que les ratios d'autonomie financière baisseraient par rapport à leur niveau actuel. Le point qu'a relevé la commission des finances concerne les conséquences de cette contraction à droit constitutionnel et organique constant. Vous le savez, le fait que les ressources propres doivent obligatoirement représenter une part déterminante de l'ensemble des ressources des collectivités territoriales imposerait de prendre rapidement des mesures correctives. Pour parler simplement, il faudrait « reterritorialiser » des impôts nationaux ou créer de nouveaux impôts locaux, pour un montant de l'ordre de 35 milliards d'euros, une fois achevées la réforme de la taxe d'habitation et une éventuelle réforme des impôts de production, si cette

Est-ce à dire qu'il faut rejeter cette nouvelle définition des ressources propres et ne jamais envisager de renforcer le pouvoir fiscal des collectivités territoriales ? Non, bien sûr ! Cela nous appelle en revanche à nous interroger sur le bon niveau de ressources propres que nous souhaitons prescrire et à préparer la réforme de la péréquation. Sur ce point, la commission des finances est satisfaite de la décision de la commission des lois de proposer que les ressources propres représentent une part significative, et non plus déterminante, de l'ensemble des ressources des collectivités territoriales. Cette part devrait-elle être de 50 % ou de 33 % ? Devrait-elle être la même pour les différentes catégories de collectivités ? Faut-il même, d'ailleurs, retenir un niveau plancher ou mettre en miroir des ressources et des charges ? La rédaction proposée ouvre le champ pour ce débat,

les textes qui nous sont proposés répondent pleinement, s'agissant de la question des compensations et des ressources propres, aux attentes de la commission des finances ; je vous invite, par conséquent, à adopter sans réserve l'article 5 de la proposition de loi constitutionnelle

je me réjouis d'être avec vous aujourd'hui pour évoquer ces deux textes, intitulés « Pour le plein exercice des libertés locales », dont je vous remercie. Ces derniers mois, au sein de la chambre des territoires, nous avons eu l'occasion d'échanger à plusieurs reprises sur la décentralisation, avec, chaque fois, de riches échanges qui nous permettent d'aller plus loin dans la nouvelle donne territoriale que nous mettons en oeuvre pour le pays. La décentralisation, vous le savez, est en effet au coeur des réflexions du Gouvernement, nous en avons encore parlé ce matin lors de la rencontre entre l'État et les collectivités locales présidée par le Premier ministre en présence du président du Sénat. L'an dernier, à l'issue du grand débat national, le Président de la République m'avait chargée de proposer un nouveau texte sur le sujet, ou, pour être tout à fait précise, sur l'évolution du cadre de relations entre l'État et les collectivités territoriales. L'objectif était clair et nous n'en avons pas dévié depuis : répondre au double besoin, très clairement exprimé par les élus et nos concitoyens, de proximité et d'efficacité des politiques publiques. C'est la raison pour laquelle j'ai lancé, le 6 janvier dernier, à Arras, une série de concertations régionales pour recueillir sentiments, réflexions et propositions de l'ensemble des acteurs de terrain, à commencer par les élus locaux. Dans ce cadre, si la crise sanitaire a perturbé le calendrier prévu, elle a aussi confirmé notre volonté initiale de donner plus de liberté aux collectivités- je note déjà un point de convergence sémantique -, notamment au regard de la réelle capacité d'adaptation et d'action dont celles-ci ont su faire preuve ces derniers mois, et ce, d'autant plus que le plan de relance leur confère une place majeure. Très bien ! Après ces mois de réflexions et de travaux, cette vision va se concrétiser prochainement au sein de deux textes dont vous avez déjà largement entendu parler. Le 29 juillet, après validation par le Conseil d'État, j'ai présenté un projet de loi organique au conseil des ministres pour assouplir les expérimentations territoriales prévues à l'article 72 de la Constitution. S'agissant du projet de loi ordinaire, il viendra consacrer les trois principes de décentralisation, de différenciation et de déconcentration-

ce fameux projet de loi dit « 3D » soit présenté en conseil des ministres en janvier 2021 et qu'il soit examiné au cours du premier semestre. Je poursuis en ce sens les concertations régionales ainsi que les échanges avec les associations d'élus, notamment dans le cadre de la réunion entre l'État et les collectivités locales qui s'est tenue ce matin. Signe de la vitalité et de l'importance capitale de ces sujets pour notre pays, nous examinons ce jour deux propositions de loi constitutionnelle et organique issues des issues des recommandations formulées en juillet dernier par le groupe de travail sénatorial. Avant toute autre considération, je tiens à dire que je constate de nombreuses convergences de vues sur l'avenir de la décentralisation, ... Tant mieux ! ... en particulier pour ce qui est de donner davantage de liberté aux collectivités locales, lesquelles doivent naturellement avoir les moyens d'être encore plus dynamiques face aux nombreux défis qui les concernent,

voire de divergences, sur lesquelles je tiens à formuler quelques précisions. Pour ce qui est du projet de loi constitutionnelle, au-delà de quelques orientations, je souhaite vous faire part d'un certain nombre de réserves. Je crois d'abord, pour citer la célèbre formule de Montesquieu, que l'on ne touche à la loi, et à la Constitution, que d'une main tremblante. Il ne s'agit pas d'une opposition de principe puisque, vous le savez, le Gouvernement avait déposé un projet de révision constitutionnelle dont je regrette- comme vous, je suppose ! -qu'il n'ait pas abouti. J'observe cependant, non sans plaisir, que vous en avez repris certaines formulations. Je crois toutefois,

de la même manière, d'ailleurs, que la décentralisation. Or ces équilibres sont le fruit d'un long travail de stratification historique, de modification très lente des rapports de force, de mouvement d'ajustement plein de gravité et que, en ce domaine, la prudence, qui est, pour Aristote, la vertu qui permet de délibérer sur ce qu'il convient de faire en fonction de ce qui est bon ou mauvais, doit dominer notre conduite à tous. à tous. Sur certaines de vos propositions, j'assume pleinement de vouloir faire preuve de prudence s'agissant d'un cadre qui garantit déjà, aujourd'hui, de réelles possibilités d'adaptation. Vous souhaitez inscrire dans la Constitution le principe de représentation équitable des territoires et ainsi accroître les possibilités de dérogation au principe de représentation sur un fondement essentiellement démographique vous cherchez donc à favoriser, par exemple, une représentation plus équilibrée de toutes les communes au sein de l'intercommunalité. Cet objectif est louable et je voudrais rappeler l'historique de cette question, car, bien que je croie fortement à la force des accords locaux pour construire les intercommunalités, force est de constater que ces derniers doivent nécessairement être encadrés pour assurer une juste représentation de toutes les communes au sein de l'espace intercommunal, j'ai d'ailleurs entendu Philippe Bas le dire il y a quelques instants.

En ce qui concerne la clause générale de compétence, je voudrais vous rassurer sur le fait que le nul n'envisage de la remettre en cause.

S'agissant du principe de compensation financière des transferts de compétences ainsi que du principe d'autonomie financière des collectivités territoriales, je rappelle que notre cadre constitutionnel actuel est déjà protecteur et équilibré. Quand l'État transfère des compétences, il accorde les ressources qu'il mobilisait à cette fin à la collectivité. Bien entendu, personne ne s'attend à ce qu'il prenne à sa charge les choix ultérieurs de la collectivité ni pour compenser des décisions coûteuses ni pour lui reprendre les ressources qu'elle dégagerait par une gestion plus efficiente. Il me semble donc périlleux, voire contre-productif d'entrer dans une logique de réévaluation permanente qui serait contraire, de surcroît, au principe de responsabilité. Je rejoins en cela, en partie, la commission des finances. Quant à votre demande d'autonomie fiscale, et non financière, je suis convaincue qu'il faut en débattre. Les régions ne disposent plus d'impôts locaux ni du pouvoir de fixer je vous pose la question : diriez-vous qu'elles manquent d'autonomie ? Je n'en suis pas certaine. Eh oui ! Ce n'est pas ce qu'elles disent ! ! S'agissant de la proposition de fusion des articles 73 et 74 de la Constitution relatifs au régime constitutionnel des territoires ultramarins, vous savez qu'il s'agit d'un sujet extrêmement sensible et complexe. À mon sens, toute évolution devrait être précédée d'une étude et d'une concertation approfondie. Le Gouvernement entend le souhait des collectivités ultramarines de disposer de statuts sur mesure qui tiennent compte pleinement de leurs caractéristiques et des contraintes spécifiques qui s'imposent à elle. Toutefois l'histoire institutionnelle de la V République, et particulièrement la révision constitutionnelle de 2003,

de loi organique, je tiens à souligner la très grande proximité entre votre texte et celui que je présenterai le 3 novembre prochain, ce dont je me réjouis, tant cela nous simplifiera les choses. me semble que nous partons en effet du même principe : l'égalité devant la loi, nécessairement générale et abstraite, demande parfois à être contrebalancée par un principe d'équité, afin de permettre à l'État de prendre pleinement en compte la singularité de chacun des territoires et aux territoires d'exprimer cette singularité à travers des réflexions, des projets, des politiques qu'ils souhaitent mener. Tel était d'ailleurs le sens du propos du Président de la République lorsque, dès la première conférence des territoires, ici même, en juillet 2017, il avait souligné que l'égalité qui crée de l'uniformité n'assure plus l'égalité des chances sur la totalité de notre territoire. C'est pour C'est pour cela que nous allons consacrer le droit à l'expérimentation et à la différenciation au sein d'un projet de loi organique que nous examinerons ensemble dans deux semaines. Concrètement, nous allons faciliter l'accès aux expérimentations pour les collectivités locales, afin d'ouvrir la voie à une différenciation durable, non pour rompre l'égalité des territoires devant la loi- les garde-fous sont nombreux et puissants -, mais pour adoucir certaines rigidités parfois stérilisantes. Vous avez l'objectif de pérenniser les expérimentations sur une partie seulement du territoire ; j'y suis évidemment favorable, mais je crois que nous devons aller plus loin et faciliter aussi le processus d'entrée dans l'expérimentation. En effet, les collectivités ne sont souvent pas demandeuses de transferts généralisés de compétences, mais d'adaptations locales. Or l'expérimentation permet précisément de répondre à ce besoin il faut donc inciter les collectivités territoriales à y recourir en simplifiant les procédures, par exemple en supprimant le rapport annuel du Gouvernement, mais pas le reste.

afin de décider s'il convient de la pérenniser sur tout ou partie du territoire ou de l'abandonner. C'est pourquoi je propose de maintenir la borne de cinq ans prévue aujourd'hui par notre Constitution. Tel est l'objet du second amendement du Gouvernement, le premier concernant les procédures. Vous le savez, cette nouvelle étape de la décentralisation sera concrétisée par le projet de loi 3D que je porte, je porte, au premier semestre de l'année prochaine, puisque ce dernier hébergera les premières expérimentations lancées sur la base du nouveau corpus que nous allons bâtir ensemble. Depuis 2017, nous agissons pour, partout, débrider les initiatives et les projets des collectivités territoriales qui inventent, au quotidien, l'avenir de notre pays.

parce qu'ils reposent sur des principes clés qui guident notre action depuis plus de trois ans, c'est-à-dire la confiance et la liberté, et donnent de nouveaux moyens concrets pour imaginer et pour mettre en oeuvre les milliers de projets et d'initiatives qui, sans cela, n'auraient peut-être pas vu le jour. La parole

Cette ambition, réaffirmée par le président Gérard Larcher, nous la partageons, ainsi qu'en a témoigné notre proposition de résolution pour une nouvelle ère de la décentralisation adoptée par le Sénat au mois de juin. Il semble que le Premier ministre la partage également, au moins dans les discours. Faisant preuve d'un jacobinisme absolu au service d'un libéralisme assumé, l'exécutif, à chaque crise, tend à se rendre progressivement compte du rôle des collectivités locales et de l'impasse de la verticalité crise des « gilets jaunes », crise sanitaire et, désormais, menace terroriste. Pointant hier cette double crise, le Premier ministre en appelait à « travailler de concert » pour combattre le terrorisme et engager une relance « ancrée dans les territoires quelle décentralisation souhaitons-nous pour que la République tienne toutes ses promesses et ne perde aucun territoire ? Quelle décentralisation souhaitons-nous pour remettre le service public au coeur de nos politiques publiques locales et redonner confiance aux citoyens ? Quelle décentralisation souhaitons-nous pour une « République jusqu'au bout » ? C'est une des questions que pose une actualité sidérante à maints égards. Si nous partageons une culture commune des territoires, nous avons cependant une différence d'appréciation globale : le texte fait le « pari de la liberté

En d'autres termes, le territoire ne peut être le lieu de la guerre de tous contre tous. Notre groupe est plus attaché aux principes d'égalité- qui ne signifie pas uniformité -et de fraternité entre les territoires qui nous a sans doute collectivement fait défaut. C'est, en tout état de cause, la condition du juste équilibre de l'aménagement du territoire. S'agissant des deux textes que nous examinons aujourd'hui, nous nous rejoignons sur plusieurs points la constitutionnalisation de la clause de compétence générale des communes par une reprise de la loi de 1884, l'assouplissement des modalités de l'expérimentation, la différenciation des compétences- sur ce point, la rédaction issue de la commission nous semble plus opportune et plus conforme à l'avis du Conseil d'État -, la différenciation normative-

à l'oeuvre depuis 2017 la suppression de la taxe d'habitation et, désormais, d'une partie des impôts de production. En revanche,

Certes, la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur la représentativité est trop limitative ; toutefois, l'inscription d'un « tunnel » de 50 % pour les EPCI nous semble excessive. Il n'est pas possible que l'avis que l'avis d'un élu puisse avoir le poids de celui de trois autres ; cela reviendrait à déséquilibrer complètement le fonctionnement des conseils communautaires.

Nous considérons également que la prise en compte de l'intérêt général est importante. Nous proposons, pour le symbole, une loi de financement des collectivités territoriales,

de nouveaux indicateurs dans les études d'impact, parce qu'il faut en finir avec le fétichisme du PIB.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, bien que j'aie pu intervenir à plusieurs reprises depuis le début de mon nouveau mandat, qu'il me

partagé, j'en suis sûr ! -de m'exprimer ici ce jour pour rappeler que, si cette confiance m'a été accordée, c'est parce qu'elle repose

Les communes sont, comme l'a rappelé le président de notre illustre assemblée, le socle de notre République. J'ajoute qu'elles constituent le quotidien de chaque citoyen. La proposition de loi qui vise à graver dans le marbre de la Constitution la clause générale de compétence et la libre autonomie des communes est frappée au coin du bon sens, car les communes ne fonctionnent que par et pour le bon sens, l'efficacité au service quotidien des citoyens. Elles reposent sur les réalités, aux antipodes de l'action du Gouvernement. S'il fallait s'en convaincre, durant la crise du covid du mois de mars, les conséquences de l'impréparation et de l'incompétence l'incompétence du Gouvernement ont été atténuées par les initiatives des maires. Heureusement que ceux-ci et leurs adjoints étaient sur le terrain pour protéger leur population. Comme il ne suffit toujours pas

particulier quand l'État réduit ses dotations financières, réveillant un autre atavisme centralisateur, celui des métropoles ? Je vous mets en garde, mes chers collègues, contre ce nouveau jacobinisme incarné par les métropoles. Rendons la liberté aux mairies et aux communes, à condition de leur en donner les moyens financiers et les prérogatives pour fonctionner au service de nos concitoyens. Hors sujet

depuis plusieurs mois, la situation liée à la pandémie de covid-19 nous permet d'apprécier la réactivité et l'étendue des actions menées sur le terrain, au service des citoyens, par les collectivités locales. Or depuis plusieurs années, force est de constater une tendance inacceptable à la recentralisation. Cette évolution s'observe d'abord au niveau financier, par un contrôle intrusif exercé sur les dépenses de fonctionnement des collectivités territoriales, mais également par l'assèchement de leurs ressources, notamment la suppression de la taxe d'habitation. Cette évolution se vérifie également au niveau normatif. La liberté des collectivités territoriales est mise à mal par un nombre excessif de normes réglementaires, l'initiative locale se traduisant par la seule mise en oeuvre de politiques nationales.

Elles visent à donner un nouvel élan aux libertés locales et à consacrer leur reconnaissance. Ces deux textes visent ainsi quatre objectifs : la représentation équitable des territoires, l'adaptation des compétences des collectivités aux réalités locales, la garantie de l'autonomie financière des collectivités et la réforme du statut constitutionnel des territoires ultramarins.

je me réjouis qu'à la formulation initialement proposée, qui visait à clarifier le contenu effectif de la clause de compétence générale, elle ait préféré la formulation traditionnelle de cette clause, selon laquelle le conseil municipal « règle par ses délibérations les affaires de la commune

dont l'exercice est attribué aux collectivités locales, selon le principe « qui décide paie ». Je rejoins la position de la commission des lois, qui a apporté plusieurs modifications tirant ainsi les conclusions du choix opéré sur la redéfinition des ressources propres en inscrivant la notion de « part significative des ressources totales » à l'article 72-2 de la Constitution. Elle a également remplacé la notion de « réévaluation régulière » par celle de « réexamen régulier », afin que la mise en oeuvre du dispositif permette d'envisager, à terme, une renégociation concertée et une révision de la gouvernance des finances locales. Enfin, elle a précisé le dispositif de compensation financière pour qu'il ne s'applique qu'aux seules modifications des conditions d'exercice des compétences de ces collectivités territoriales résultant de décisions de l'État. Le troisième et dernier point que je souhaite aborder porte sur la nécessité de rénover le régime constitutionnel des collectivités d'outre-mer. Afin que ces dernières disposent d'un cadre constitutionnel plus souple, qui permette d'adapter davantage leurs institutions aux réalités locales, l'article 6 de la proposition de loi constitutionnelle prévoit de fusionner les articles 73 et 74 de la Constitution. Je me félicite tout particulièrement de ce que la commission des lois ait considéré que le contenu de cet article était équilibré. Madame la ministre, mes chers collègues, partageant pleinement les objectifs visés par ces deux propositions de loi, le groupe Les Indépendants, particulièrement attaché au maintien des libertés locales au coeur de notre organisation administrative, votera ces textes.

en attestent-sont le bon levier pour agir en proximité. La crise sanitaire a d'ailleurs montré le rôle essentiel des collectivités pour agir dans l'urgence et apporter les réponses adaptées aux attentes et aux besoins de la population.

continuer longuement. Nous pensons que le renouvellement de notre démocratie locale ne figure pas dans ce texte. Nous estimons que la coopération territoriale et le recours à la contractualisation pour renforcer la réciprocité entre territoires urbains et ruraux auraient dû faire l'objet

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous statuons, cet après-midi et ce soir, sur l'initiative de groupes politiques qui entendent apporter un accroissement, d'ailleurs plutôt volumineux, à la Constitution sur le champ des relations entre l'État et les collectivités territoriales, relations que ces groupes se donnent pour objectif de transformer en profondeur.

qui, de manière beaucoup plus sobre, a établi deux principes qui ont leur place dans la Constitution : celui de la République décentralisée et celui de la garantie des ressources financières des collectivités territoriales.

un article 72-1 avait alors été introduit dans la Constitution pour permettre l'organisation de votes directs des citoyens -votes indicatifs ou délibératifs suivant les cas.

Nous pensons donc nous positionner de façon défavorable à cette proposition de loi constitutionnelle, et cela en raison de deux objections majeures.

Je rappelle d'ailleurs à ceux qui font reproche au Conseil constitutionnel d'avoir établi une relation chiffrée de 1 à 1,5, c'est-à-dire de 80 % de la moyenne à 120 % de la moyenne de population représentée, que cette disposition a été adoptée dans les deux assemblées lors de la révision des circonscriptions en 2009. Tout le monde a alors trouvé naturel de limiter à un écart de 1 à 1,5 le pouvoir de vote et le pouvoir de participation à la délibération générale entre deux citoyens.

la volonté d'affaiblir, voire, en creux, d'abolir le pouvoir de l'État en matière de régulation des services publics lorsqu'ils donnent lieu à des transferts de compétences. L'idée de priver l'exécutif de son pouvoir réglementaire d'application de la loi lorsqu'il tend à régir des compétences qui ont été décentralisées, en oubliant que ces mêmes compétences consistent à exercer des services publics à assurer des missions d'intérêt public au service des citoyens, cette idée de priver l'exécutif du pouvoir d'établir des normes générales qui sont des garanties d'égalité entre les citoyens

la pensée éthérée et constitutionnelle, et que nous devons nous opposer à ces excès. En revanche, comme l'a dit Mme la ministre, la proposition de loi organique, elle, établit un schéma de déroulement et de conclusion des expérimentations qui se rapproche du travail

vaste projet pour nous que de vouloir garantir le plein exercice des libertés locales ! Vaste projet, car les vagues de décentralisation se sont succédé, les transferts de compétences également, mais les moyens financiers, eux, se sont souvent réduits. En parallèle, le rôle des élus a lui aussi évolué-je pense en particulier aux maires de petites ou très petites communes comme il en existe beaucoup chez moi, en Lozère. D'abord, la montée de l'individualisme a profondément changé le rapport maire-administrés. Loin de la figure tutélaire, le maire est souvent désigné comme le premier responsable des dysfonctionnements face à des administrés toujours plus exigeants. Ensuite, l'inflation législative a créé de nombreuses contraintes pour nos territoires : ils n'ont souvent ni les moyens financiers ni l'ingénierie nécessaires pour y faire face. Dernière évolution, et non des moindres, l'intercommunalité, qui, si elle peut être un formidable catalyseur à l'échelon local, a aussi ses failles-nous les connaissons. La principale est la faible représentation des petites communes, qui fait que certaines d'entre elles, faute d'être considérées, se désintéressent du fait intercommunal, voire s'y opposent frontalement.

Concernant les dispositions visant à garantir une représentation équitable des territoires, notre groupe, comme en 2014, est pleinement favorable à la constitutionnalisation de ce principe. Sa mise en oeuvre concrète, par la hausse des limites maximales d'écart de représentation, est une avancée appelée depuis de nombreuses années par les élus des petites communes et par le RDSE. Nous ne pouvons donc qu'y être favorables. Couplée à cette mesure, la clause générale de compétence vient rappeler l'importance de la commune dans l'édifice juridique français. S'agissant de l'adaptation des compétences des collectivités aux réalités locales, nous sommes favorables aux dispositions de l'article 2 de la proposition de loi constitutionnelle, qui permet de clarifier l'exercice du pouvoir réglementaire local. Cet article s'inscrit dans la droite ligne du principe de libre administration des collectivités reconnu par l'article 72 de notre constitution. Cet ajout permettra la différenciation prévue à l'article 3. L'octroi de compétences distinctes à des collectivités locales de même échelon, s'il peut parfois s'avérer nécessaire, doit rester calibré pour être efficace. Notre crainte est une différenciation sans borne qui conduirait à une disparition progressive des trois échelons que sont la région, le département et la commune. Or force est de constater que cette version ne nous satisfait pas l'alinéa 8 de l'article 3 de la proposition de loi constitutionnelle renvoie à une future loi organique, mais ne donne pas de cap. Plus globalement, la méthode employée nous dérange. Personne ici n'est sans savoir que le projet de loi 3D sera prochainement examiné. C'est pourquoi l'examen de ce texte, inscrit à l'ordre du jour il y a quelques semaines seulement, nous interroge. Non pas que le Sénat ne devrait plus prendre d'initiatives- loin de là mais, sur ces sujets de grande importance, tâchons de travailler en bonne intelligence pour établir un texte à la hauteur des attentes des élus locaux. Pour en revenir aux textes que nous examinons, je rappelle que le RDSE a toujours été favorable à l'autonomie fiscale et financière des collectivités locales,

Nous craignons que l'autonomie que vous proposez ne débouche sur une mise à mal de la péréquation, avec des communes riches qui vont devenir toujours plus riches et des communes pauvres qui vont l'être encore plus. Élue d'un département hyper-rural, ces questions me touchent tout particulièrement ; c'est pour cela que j'en appelle à votre vigilance. On me répondra que les transferts de compétences sont compensés intégralement à date de ces transferts,

Si nous sommes naturellement favorables aux mesures visant à consacrer une représentation équitable des territoires, nous avons des craintes quant à vos conceptions de la différenciation et de l'autonomie fiscale et financière des collectivités territoriales.

les principes de libre administration et d'autonomie financière des collectivités ont été méprisés par les gouvernements. La réforme de la taxe d'habitation, puis la baisse de la fiscalité économique locale proposée dans le projet de loi de finances pour 2021 se situent malheureusement dans cette droite ligne. Les élus locaux sont à bout face à l'érosion de leurs marges de manoeuvre et face au comportement autoritaire du Gouvernement, qui leur impose cette austérité budgétaire.

Cette clause de compétence assure aux élus locaux de l'espace, de la liberté pour innover, adapter sur le terrain tout en restant dans le cadre républicain de l'égalité des citoyens devant la loi. monsieur Ravier, la loi est la même pour tous et partout en République. Cela ne remet pas en cause la libre administration des collectivités territoriales, mais garantit à chacune et à chacun, quelle que soit sa condition sociale et territoriale, d'être un citoyen de la République. Je note d'ailleurs que M. Ravier, bien que passionné par les collectivités territoriales, nous a déjà quittés Indissociable de la liberté locale, l'autonomie financière est le levier d'action des élus : sans finances, il n'y a pas de compétences. Les coupes dans les ressources propres sont depuis trop longtemps dissimulées de manière artificielle par le remplacement d'impôts locaux avec un pouvoir de taux par des compensations et transferts de parts d'impôts nationaux. Nous évoluons vers une fiscalité locale recentralisée, qui est non plus un outil budgétaire dans les mains des élus, mais un outil d'assujettissement du Gouvernement. Sans capacité d'action locale ni maîtrise des ressources financières, le lien entre citoyens et élus locaux s'étiole, et la démocratie locale, vidée de toute concrétisation,

à chacun sa définition, certes, mais il nous faudra en avoir une définition commune. La crise actuelle a créé une tension inévitable et incontestable entre le local et le national. L'action et la communication gouvernementales ont beaucoup déçu. De nombreux élus et citoyens se sont retrouvés démunis, encore aujourd'hui, madame la ministre, face à l'absence de concertation pour l'instauration du couvre-feu. Des velléités d'indépendance accrue ont donc pu se développer dans ce climat prônant un pouvoir local plus apte que le national à réagir. C'est souvent vrai, mais de telles demandes peuvent aussi se trouver mêlées aux désirs et particularismes locaux qui menacent le cadre républicain d'unicité et d'indivisibilité de la France, d'où le besoin de plus de décentralisation, mais aussi de plus de République, de plus de déconcentration pour sécuriser l'action des élus locaux. C'est dans ce contexte que vous proposez d'introduire les concepts de représentation équitable des territoires et de différenciation territoriale. Les débats à ces sujets sont légitimes et doivent nourrir notre réflexion. La différenciation que vous proposez de développer par l'attribution de compétences différentes aux collectivités

pour les citoyens. Il y a donc de réels risques de ne plus contrôler ce que la différenciation créera. En cette période compliquée, la prudence nous semble donc être le maître mot. C'est pourquoi, en l'état, le groupe CRCE votera certains articles, mais il ne votera pas ces propositions de

sur ces travées, depuis toujours, nous veillons à l'autonomie et au respect de nos collectivités. Nous veillons à ce que leurs dotations ne baissent pas et à ce que les élus soient reconnus. Pour autant, nous n'avons pas toujours été entendus, en particulier lors du débat sur la loi NOTRe, loi que beaucoup aujourd'hui considèrent comme funeste.

Il me paraît donc que le moment est à saisir pour repenser, adapter, voire alléger le fonctionnement de nos collectivités. Tel était l'objectif de la délégation aux collectivités territoriales

assurer une représentation équitable des collectivités, adapter leurs compétences à leur réalité, garantir leur autonomie financière et, enfin, réviser le régime constitutionnel de nos collectivités ultramarines. Une représentation

Combien de communautés de communes ou de communautés d'agglomération dysfonctionnent-elles, parce que les plus petites communes n'ont plus voix au chapitre et que la ville-centre, majoritaire à elle seule, gère l'agglomération comme si c'était chez elle, et uniquement chez elle ? Et je ne parle pas de la métropole de Lyon au sein de laquelle certaines communes ne sont plus représentées, niées, trop petites, alors que le confinement nous a prouvé la véritable utilité des petites communes. Parlons des compétences, maintenant. Ces textes permettront une adaptation des compétences en fonction de ce que les collectivités peuvent, veulent ou non réaliser. Il me semble que c'est le volet le plus difficile à mettre en oeuvre. le fait de permettre à une collectivité d'exercer une mission qu'elle souhaite exercer alors que, dans la collectivité voisine, c'est à un autre échelon que l'affaire se traite, à créer de l'inégalité. Mais doit-on empêcher une commune de réaliser une action qui relève du ressort communautaire si l'EPCI ne s'en saisit pas ? Les communes en question, me direz-vous, disposent peut-être de moyens que les autres n'ont pas. Mais peut-être veulent-elles justement mettre les moyens que d'autres ne souhaitent pas y consacrer. Et peut-être est-ce cela justement faire de la politique ? C'est pourquoi il est bon de voir un texte limitant le pouvoir réglementaire national sur les collectivités, tout comme il est bon de constitutionnaliser la clause de compétence générale des communes. Alors, c'est vrai, il n'y aura pas les mêmes avantages à vivre dans la collectivité X que dans la collectivité Y, mais c'est à cela que servent les élections : choisir ses élus et son cadre de vie. dans la proposition de loi organique des études d'impact et des avis du Conseil national d'évaluation des normes, ainsi que la possibilité introduite par nos collègues socialistes de faire appel à des organismes publics indépendants pour réaliser ces études d'impact. Toujours parmi les sujets de satisfaction, j'ajoute l'allongement de la période d'expérimentation et la possibilité, au terme des expérimentations, de les étendre à tout ou partie- et c'est bien entendu le mot « partie » qui m'intéresse -du territoire. les ressources, ensuite. Comment ne pas approuver que celles-ci puissent être déconnectées des impôts nationaux, sur lesquels les collectivités n'ont aucune prise ? Par ailleurs, on nous retire la taxe d'habitation, coupant ainsi un lien fort- quand bien même n'est-il pas agréable -entre la commune et ses habitants. Tailler dans les ressources propres des communes revient à mettre ces dernières sous tutelle, car on les rend ainsi dépendantes des dotations. Comment définir une politique si l'on ne peut définir les moyens à y consacrer ? Je comprends donc cette dissociation même si, là encore, je crains que nous n'attendions longtemps avant que celle-ci puisse s'appliquer. revanche, et cela devrait être mis en place rapidement, il est indispensable de prévoir le réexamen régulier des moyens affectés aux politiques décentralisées.

Cela doit nous servir d'exemple, afin que nous n'acceptions pas une nouvelle décentralisation- quand bien même serait-elle souhaitée -sans compensation financière et sans clause de réexamen régulier. les collectivités ultramarines, enfin. Notre groupe compte des élus ultramarins, qui ont su nous sensibiliser à leurs problèmes. Notre collègue Lana Tetuanui a proposé plusieurs amendements, qui ont été rejetés par la commission. Ils visaient à aider la collectivité de Polynésie- mais les difficultés rencontrées par les uns doivent l'être par les autres -à mieux s'administrer. Pour autant, dans sa sagesse, la commission a limité l'intervention de ces propositions de loi sur les articles 73 et 74 de la Constitution, ouvrant le débat, mais préférant laisser mûrir les sujets avant de les faire entrer dans la loi. je rappelle que toutes nos collectivités- je dis bien « toutes » -, si proches ou lointaines soient-elles de Paris, ont besoin de souplesse et de réactivité de la part de l'État. Toutes ont besoin de bon sens et d'agilité.

confiance, proximité, autonomie, ce sont davantage que trois mots : ce sont les socles des libertés locales, les bases d'une gestion locale à la hauteur des attentes de nos concitoyens, les fondements de la cohésion nationale tant ébréchée aujourd'hui. La représentativité est en crise : face au besoin de proximité, c'est encore le sentiment d'éloignement qui règne aujourd'hui. La crise des gilets jaunes a mis en exergue le sentiment d'abandon dans nos territoires et dans notre réalité.

nos concitoyens retrouveront le chemin des urnes lorsqu'ils auront le sentiment que les décideurs, les élus, l'administration apportent des solutions à leurs préoccupations dans une démarche sincère, désintéressée et efficace. À cela s'ajoute le trop-plein de normes générales, édictées d'en haut. L'horizontalité de la prise de décision doit succéder à la verticalité. Comme le met en valeur la présente proposition de loi constitutionnelle, doivent désormais succéder une décentralisation plus approfondie et la confiance en nos élus locaux : ces derniers ont la connaissance et l'expérience du terrain que ne possède pas le pouvoir central. Cette étape nécessaire permettra de retrouver la proximité. Le principe de subsidiarité devrait être appliqué face à la logique réglementaire centralisée, qui domine en France. Aussi, la territorialisation des politiques publiques doit aujourd'hui devenir un impératif.

et cette demande est légitime : c'est la base de la cohésion nationale, de l'équité territoriale et des libertés locales. La crise sanitaire a une fois de plus la responsabilité, la capacité à réagir et à gérer, l'exemplarité de nos collectivités locales, de nos communes, pour faire face à une situation urgente et assurer une gestion au quotidien dans l'inconnu. Celles-ci ont fait preuve de réactivité, alors qu'elles avaient été honteusement balancées auparavant avec le hashtag #BalanceTonMaire. La clause générale de compétence de nos communes doit donc assurément être consacrée dans la Constitution. Nos communes ont largement fait leurs preuves et ont, une fois de plus, été au front : après la première ligne des soignants, nos maires et nos élus locaux étaient en deuxième ligne. Elles doivent donc garder les moyens de leur action sur le moyen et le long terme. L'État doit leur faire confiance, mais, la confiance, cela ne se décrète pas : cela se vit au jour le jour, dans l'exercice des fonctions et dans la facilité accordée à la résolution des problématiques. Ces propositions de loi sont l'occasion pour l'État de montrer sa confiance aux élus locaux. Vous devez saisir cette opportunité, madame la ministre, pour renouer le lien avec nos collectivités locales, nos communes, nos territoires. Renouer le lien, c'est aussi renouer avec la proximité telle que l'affirmait la proposition de loi organique visant à garantir une République de proximité de notre collègue Rémy Pointereau, qui prévoyait très justement la possibilité d'exercer de manière concomitante un mandat de parlementaire et celui de maire d'une commune de moins de 9 000 habitants ou celui de président d'une intercommunalité de moins de 15 000 habitants. Des parlementaires déconnectés du terrain, on en voit depuis trois ans ! Ils n'ont pas véritablement fait leurs preuves La suppression de la réserve parlementaire est allée dans le même sens : elle est révélatrice d'un État jacobin, qui donne du pouvoir aux représentants de l'État et l'enlève aux élus de terrain. Or nos édiles locaux portent la légitimité à élaborer et à soutenir des projets de territoire. Enfin, qu'on le redise à l'occasion de l'examen de cette brillante proposition de loi constitutionnelle : la liberté passe par l'autonomie et, notamment, l'autonomie financière. La pratique actuelle va à l'encontre de celle-ci, à l'exemple de la suppression de la taxe d'habitation par l'État, sans pour autant que la ressource supprimée soit suffisamment compensée. Il s'agit d'une atteinte claire à la liberté d'action de nos collectivités locales : c'est inacceptable ! Cela va à l'encontre de la demande de démocratie locale de nos concitoyens. Cela va à l'encontre de la demande de davantage de proximité. Pour conclure, mes chers collègues, madame la ministre, je dirai tout simplement : arrêtons de faire de l'aménagement du territoire et faisons de l'aménagement territoires ! Il me semble essentiel d'affirmer que, pour nous élus, la décentralisation ne peut que s'effectuer et se vivre dans la confiance, la proximité et l'autonomie.

la démarche engagée par le groupe majoritaire pour plus de territorialisation, plus de différenciation, plus de stabilité financière et plus de sécurisation juridique, même si nous récusons le seul prisme de la liberté territoriale. Sur ces travées, ces travées, nous n'avons pas peur des libertés locales. Nous convenons aussi qu'il est désormais nécessaire de faire respirer la Constitution pour permettre à chaque territoire de s'épanouir au sein de notre République. Depuis trop longtemps, ici, dans l'Hexagone, mais aussi dans tous les territoires d'outre-mer- ou presque -, nous attendons une évolution de notre Constitution. Chacun voit bien ici, bien loin des slogans trop longtemps martelés, que l'« uniformisme » des politiques nationales demeure trop souvent la règle, et la différenciation un mirage. En résultent des politiques publiques parfois déconnectées de nos réalités et peu efficaces pour nos populations. Pour être tout à fait honnête, nous autres élus en prenons toute notre part. Il faut résolument avancer vers plus de pouvoir décisionnel local, vers un échelon local doté de réels pouvoirs normatifs, tout en réaffirmant l'unité de la République : telle est la ligne de crête.

qui doit inéluctablement être fait par les populations et les peuples, les parlementaires que nous sommes ne peuvent se défiler devant leurs responsabilités.

Il s'agit ici d'affirmer notre volonté de cranter des avancées et des convergences de pensée. Nous sommes tous farouchement attachés aux principes de liberté et d'égalité, et non d'égalitarisme. Dans les outre-mer, leur concrétisation devra tôt ou tard passer par une réforme constitutionnelle. Depuis plusieurs années, chacun chemine à sa façon et à son rythme. Jusqu'à présent, aucun constitutionnaliste n'avait proposé un dépassement de la logique binaire entre spécialité et identité législative, incarnée par les articles 73 et 74 de la Constitution. Nous aurons tout à l'heure à nous prononcer sur une nouvelle rédaction que j'ose qualifier d'« efficace » et d'« ambitieuse ». C'est bien la première fois que nous avons devant nous une proposition, certes perfectible- et je pourrais y revenir -, mais pour le moins concrète et répondant, pour une grande part, à la volonté de différenciation des décideurs locaux. Par deux fois, les élus du congrès de Guadeloupe nous ont mandatés pour suivre cette affaire au niveau national.

devant la multiplicité des thèmes abordés dans ces propositions de loi et au regard de l'actuel état financier dans lequel se trouvent plongées nos collectivités, permettez-moi en cinq minutes de concentrer mon propos sur ce seul aspect budgétaire. En effet, les marges de manoeuvre financières des collectivités territoriales connaissent depuis plusieurs années une réduction sans précédent. Du côté des dépenses, les contrats dits de Cahors ont eu pour effet de contraindre très significativement leurs choix de gestion, en exerçant une forte pression à la baisse sur leurs dépenses réelles de fonctionnement. Du côté des recettes, la réforme en cours de la taxe d'habitation entérine le mouvement- déjà entamé -d'une réduction du pouvoir fiscal des collectivités au profit du transfert d'impositions nationales sur lesquelles les collectivités n'ont jamais la main. Nous sommes là bien loin de l'article 72 de notre Constitution, qui prévoit pourtant clairement que nos collectivités s'administrent librement et qu'aucune d'entre elles ne peut exercer une tutelle sur une autre. Il convient donc de remédier aux différentes dérives constatées ici ou là, en renforçant les outils de leur autonomie financière. Garantir l'autonomie financière des collectivités locales, c'est d'abord redéfinir la notion de ressources propres c'est l'objet de l'article 4 de la proposition de loi organique, qui vise à en exclure les ressources sur lesquelles les collectivités n'ont aucun pouvoir ni de taux ni d'assiette, et qui donnent une image tronquée de la réalité de leur autonomie financière. Cette redéfinition pose néanmoins des difficultés techniques, tenant au niveau des ratios d'autonomie financière qui en résultent. Nettement diminués, ceux-ci seraient surtout très inégaux, posant la question de la cohérence juridique de la notion de « part déterminante de ressources totales », qui doivent représenter les ressources propres d'une catégorie de collectivités. La commission des lois a donc choisi de remédier à cette difficulté en adoptant un amendement, pour prévoir que les ressources propres ne constituent qu'une part significative des ressources totales d'une catégorie de collectivités. Si ce choix revient à diminuer la portée de l'exigence constitutionnelle, il permet en réalité d'en garantir l'applicabilité. La commission des lois a également supprimé la procédure de modification du calcul prévu au dernier alinéa de l'article 4 de la proposition de loi organique. Celle-ci ne semblait pas répondre à une nécessité réelle, dans la mesure où l'éventuelle diminution des concours financiers de l'État s'opère généralement en dehors de toute référence au ratio d'autonomie financière et pouvait ainsi mener à l'insincérité de l'indicateur.

L'article 5 de la proposition de loi constitutionnelle vise, à titre principal, à garantir la pleine compensation financière des compétences dont l'exercice est attribué aux collectivités territoriales selon le principe « qui décide paie ». Il étend la règle de compensation financière intégrale actuellement applicable aux transferts de compétences, aux créations et extensions, mais également aux modifications des conditions d'exercice des compétences des collectivités territoriales. Il prévoit également une réévaluation régulière des ressources ainsi transférées aux collectivités. La commission des lois a adopté cet article en lui apportant trois modifications. Premièrement, elle a tiré les conclusions du choix opéré sur la redéfinition des ressources propres en inscrivant la notion de « part significative des ressources totales » à l'article 72-2 de la Constitution. Deuxièmement, elle a remplacé la notion de « réévaluation régulière » par celle de « réexamen régulier », afin que la mise en oeuvre du dispositif permette d'envisager, à terme, une refonte de la gouvernance des finances locales. elle a précisé le dispositif de compensation financière pour qu'il ne s'applique qu'aux seules modifications des conditions d'exercice des compétences des collectivités territoriales résultant de décisions de l'État. Pour conclure, à l'heure où tout le monde brandit la décentralisation telle une marotte, je précise que ces propositions de loi ont le grand mérite de placer le sujet de l'autonomie financière des collectivités au centre des débats, et c'est heureux

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nul n'ignore ici combien la différenciation territoriale est placée au coeur des réflexions et de la vision des outre-mer de Michel Magras, notamment en tant que levier du dénouement du noeud gordien de l'inadaptation des normes- au sens large -si dommageable aux territoires. Aussi, j'ai l'honneur à la fois de succéder à Michel Magras au sein de la Haute Assemblée, et d'admettre et d'assumer d'être son ombre portée dans ce débat. L'enjeu de l'acclimatation est crucial outre-mer, afin de garantir la pertinence de la norme et, ainsi, l'efficience des politiques publiques. Les travaux sur les normes de la délégation sénatoriale aux outre-mer ont en cela été fondateurs d'une nouvelle approche. C'est aussi dans cette optique que l'adoption d'un nouveau cadre constitutionnel commun aux outre-mer constitue l'aboutissement de la réflexion menée au coeur du récent rapport de la délégation, intitulé.

L'intérêt d'un tel cadre est d'offrir la possibilité de déterminer l'autorité la mieux placée pour exercer la compétence, tout en permettant à chaque territoire de définir l'organisation qui lui convient à cet effet. Dans le sillage des travaux du groupe de travail du Sénat sur la décentralisation, la majorité sénatoriale a donc souhaité examiner le présent texte dans un délai certes très court. J'y vois pour ma part une démarche de reconnaissance et d'affirmation du rôle central des collectivités, y compris outre-mer, particulièrement mis en lumière durant le confinement, et la volonté de la placer à la charnière du lien de confiance à recréer, ce à quoi on ne peut que souscrire. L'outre-mer ne saurait rester à l'écart du mouvement de desserrement de la centralisation et de renforcement de la démocratie locale qu'entend ainsi amorcer le Sénat.

même si, disons-le, cela a pu surprendre. Si cet article répond au principe de réunion des articles 73 et 74 de la Constitution, adopté par le groupe de travail sur la décentralisation du Sénat, il ne saurait pour autant occulter certaines objections sur la méthode et sur le fond. Les travaux de notre ancien collègue Michel Magras sur la différenciation territoriale ont permis d'aboutir, postérieurement au dépôt du présent texte, à une rédaction qui, sur le fond, semble recueillir une adhésion relativement large. À cet égard, la mise en place d'un groupe de travail permettrait un approfondissement de la nécessaire concertation dans le cadre bien compris des prérogatives du constituant. Je vous proposerai, par voie d'amendement, que ces travaux soient mis en oeuvre sur le fondement d'une première rédaction. La collectivité de Saint-Barthélemy n'était pas spontanément demandeuse d'une réforme en profondeur du cadre constitutionnel, mais elle considère que l'opportunité de tirer les leçons de l'expérience de son statut doit être saisie, en améliorant le cadre constitutionnel qui lui permettrait de parfaire son propre cadre statutaire. L'actuel cadre constitutionnel ne lui a, par exemple, pas permis d'être entendue sur ses aspirations en matière de sécurité sociale. Il s'agirait également de prévoir le transfert du droit pénal spécial, la procédure actuelle ayant montré ses limites.

au fond, la problématique qui nous occupe est celle de la conciliation de la pluralité des outre-mer et de leurs aspirations, qui restent malgré tout liées par leur destin constitutionnel. En dépit de trajectoires différentes, je suis convaincue que la discussion peut nous permettre de nous rejoindre.

dans le droit public local et traduit, à l'intérieur de subdivisions électorales, des circonscriptions ou des collectivités territoriales particulières et, donc,

cet écart de 400 habitants signifie que, dans une même assemblée, l'élu de la circonscription la plus peuplée représente 50 % d'électeurs de plus que celui de la commune la moins peuplée. Si nous élargissons le tunnel à plus ou moins 33 %, deux élus d'une même assemblée pourront représenter, pour l'un, 670 habitants et, pour l'autre, 1 330 Cela signifie que l'élu de la circonscription la plus peuplée représenterait une population deux fois plus importante que l'élu de la circonscription la moins peuplée. Dit autrement, un citoyen de la plus petite municipalité pèserait deux fois plus qu'un citoyen de la plus grande circonscription dans des décisions qui s'appliqueraient à chacun d'eux de la même manière. Ce sont des écarts

Avec cette disposition constitutionnelle, on prive les gouvernements, à l'avenir, d'exercer leur mission élémentaire

ne détermine que les modalités d'attribution des aides. J'ai pu constater dans un domaine extrêmement sensible, celui de l'attribution du RSA, les excès de dispositions réglementaires s'imposant aux départements.

à admettre que les départements puissent mettre en oeuvre leur propre réglementation pour l'appréciation du patrimoine à prendre en compte. Voilà un exemple concret ! Il est très important, selon moi, que le pouvoir réglementaire national soit supplétif,

C'est ainsi que le Conseil constitutionnel a admis des dérogations, qui permettent, par exemple, à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon et ses 6 000 habitants d'avoir un sénateur. Avec cet amendement, les motifs d'intérêt général pourraient être pris en compte

des communes, des élus, de leur appropriation des politiques intercommunales et, donc, des politiques menées au service des populations habitant au sein de ces intercommunalités constitue un vrai défi.

la loi Engagement et proximité a rétabli une disposition exclue par la législation antérieure.

j'ajouterai que c'est justement parce que le Conseil constitutionnel permet qu'il y ait deux représentants que votre amendement est difficile à accepter : son adoption supprimerait cette possibilité ! Enfin, je rappelle que

Je signale simplement que le Conseil constitutionnel, pour défendre le tunnel de 20 %, s'appuie sur une réflexion constante, reposant sur les limites que le législateur s'était données

eu pour effet, parallèlement à la baisse des dotations, d'encourager la création d'intercommunalités XXL, qui rendent encore plus nécessaire l'obtention d'un accord local.

de donner des marges de manoeuvre pour des accords locaux. Il me semble nécessaire, au vu des difficultés rencontrées et des remontées de toutes les associations d'élus,

Je voudrais indiquer à M. Kerrouche que je partage entièrement la position de notre corapporteur. Le sujet de l'intercommunalité, ce n'est pas l'habitant, c'est la commune Les délégués communautaires représentent la commune ! Il y a donc une différence, non pas de degré, mais de nature entre une collectivité territoriale et une intercommunalité, chargée, sur la base d'un accord entre communes, de gérer les affaires qui sont mieux gérées à son niveau qu'au niveau communal. Cela signifie, tout simplement, que nous devons créer de la souplesse. Précisément, madame la ministre, parce que le Conseil constitutionnel s'est prononcé, nous ne pouvons pas le faire autrement que par une révision de la Constitution. Cette souplesse, le législateur devra s'en emparer, du moins si cette révision est menée à son terme, de sorte que l'accord

cette campagne sénatoriale a été l'occasion de partir ou repartir à la rencontre des conseils municipaux, qui nous ont ouvert leurs portes. Chaque fois, nous y avons entendu parler de projets et avons constaté intacte cette volonté d'agir, de peser sur la vie quotidienne et l'avenir de la commune. Je l'ai moi-même constaté dans les 335 communes ardéchoises. Ces communes, elles sont le lieu de rencontre entre les modes de vie partagés, les liens humains tissés au fil des générations et la volonté d'écrire un destin commun. Elles constituent souvent le bel exercice de la démocratie, car elles permettent d'apprécier, dans la vie de chacun, les décisions prises par les élus. Sans cesse, les maires et leurs équipes doivent imaginer de nouvelles solutions et satisfaire des attentes de plus en plus impatientes. La plupart du temps, ils sont les premiers à devoir régler les problèmes du quotidien, répondre à la demande de solidarité, mais aussi réagir face aux situations de crise, qu'il s'agisse d'épidémies ou de catastrophes naturelles. Droit à l'instruction, solidarité, accès à la culture, aux loisirs, à la sécurité, à un cadre de vie agréable ... : les maires sont les maires sont des ministères de la proximité et de l'imprévu, à qui il revient chaque jour d'accomplir la promesse républicaine. Pour protéger leur capacité d'agir de la fièvre recentralisatrice qui parfois s'empare des gouvernements, il m'apparaît indispensable de la sanctuariser dans notre Constitution.

On l'a bien vu avec la crise sanitaire, les départements ont besoin de retrouver de la liberté pour répondre aux besoins de leurs habitants. Ils ont montré qu'ils étaient le bon échelon de gestion pour distribuer les masques et les équipements de protection individuelle, gérer les services départementaux d'incendie et de secours, mener une action publique de proximité. Comme l'a révélé le rapport de la mission d'information sur le rôle, la place et les compétences des départements dans les grandes régions-

l'urgence et, dans certains cas, les insuffisances de l'État ayant conduit certains départements ou certaines régions à prendre des mesures aux marges de leurs domaines d'attribution. Comme indiqué dans la synthèse du rapport, « face à de telles situations, on ne saurait se contenter d'une application des textes à géométrie variable C'est la raison pour laquelle il convient de rétablir la clause de compétence générale pour les départements, déjà reconnue en cas de catastrophe naturelle. C'est la proposition n° 16 du rapport de la mission d'information, et c'est aussi ce que demande l'Assemblée des départements de France.

Donner la compétence générale au département, c'est une nécessité. Revenir sur cette possibilité est utile pour tenir compte des caractéristiques de chaque territoire, qui doit pouvoir agir selon ses caractéristiques dans les secteurs qu'il juge le plus utiles à la fois pour lui et pour sa population, en particulier, je veux le souligner, dans le domaine économique, car c'est en proximité que l'on peut intervenir pour valoriser les ressources locales, les spécificités territoriales. spécificités territoriales. J'ai toujours eu, en tant que président du conseil départemental de 2011 à 2017, d'excellentes relations avec les différents présidents de région. Sur des projets de développement économique local, j'ai toujours eu une écoute bienveillante et généralement trouvé des solutions pour que la région accompagne ses projets de développement économique.

valeur. Effectivement, ce n'est qu'en proximité qu'on est en mesure de tirer parti des caractéristiques propres d'un territoire, que l'on est en mesure de soutenir de manière spécifique les entreprises du territoire au regard de ce qu'elles représentent et donc de ce qui les constitue. Je voudrais dire aujourd'hui : « N'ayez pas peur des départements ! » Nos concitoyens n'en ont pas peur ; ils se désolent d'ailleurs qu'on leur ait, d'une certaine manière, coupé les ailes, particulièrement dans les territoires ruraux. Les départements sont des collectivités d'avenir : permettez-leur d'agir en leur rendant cette compétence générale. La parole

Dormez en paix, braves gens, l'État pourvoit à tout ! » Il me semble quand même que la période récente, notamment la nécessité de commander en catastrophe des quantités de masques

Oui, vous avez raison, mais, ce qui intéresse encore plus les Français, c'est l'efficacité : ils veulent que ça fonctionne ! Dans certains cas, même si nous sommes tous d'accord pour sanctuariser le rôle de la commune, le département peut être plus efficace que celle-ci. Je vais vous donner un exemple très précis

Une petite commune aurait-elle eu les moyens d'apporter cette aide à ses artisans, à ses autoentrepreneurs ou autres ? Non !

Normalement, la compétence économique est dévolue aux régions, mais qui va, par exemple, faciliter la création d'une petite zone artisanale de 6 ou 8 lots dans une commune ou une communauté de communes pour permettre à l'artisan local de quitter le centre du village et de s'y

c'est de constitutionnaliser la clause de compétence générale des communes, étant entendu qu'on peut tout à fait conférer au département la clause de compétence générale sans qu'il soit pour autant nécessaire de l'inscrire dans la Constitution. Le vrai débat que nous avons à trancher ce soir, c'est celui-là

Il lui a été préféré, pour atteindre l'objectif visé d'une meilleure visibilité sur les finances locales, la création d'un débat annuel consacré aux finances locales juste avant l'examen par le Parlement du projet de loi de finances.

il nous est difficile de nous prononcer réellement sur le fond et il serait extrêmement dommageable qu'une telle disposition soit adoptée par amendement dans un véhicule qui ne me paraît pas adapté- c'est ce que je vous disais en commission alors qu'elle nécessite un travail de fond associant pleinement la commission des finances, particulièrement concernée- nous avons eu l'occasion de l'évoquer avec notre collègue rapporteur pour avis Charles Guené.

Tout d'abord, une partie des recettes locales provenant du budget de l'État, son montant ne peut donc être fixé que par une loi de finances. Je parle là des prélèvements sur recettes, en première partie de la loi de finances, et des crédits budgétaires, en seconde partie. En outre, il existerait forcément des doublons entre la loi de financement des collectivités et la loi de finances. Beaucoup de dispositions se retrouveraient dans les deux textes.

qu'il faut chevaucher le tigre. Je constate simplement que, en ce qui concerne les collectivités locales, l'audace est relativement limitée alors qu'elles mériteraient de savoir à quelle sauce elles seront mangées tous les ans.

qui leur permettrait d'exister par rapport au budget de notre pays ? C'est la raison pour laquelle nous soutenons à fond, avec beaucoup de détermination, l'amendement que vient de présenter M. Kerrouche.

vote. Je ne suis pas d'accord avec cet amendement. Monsieur Kerrouche, vous nous dites que les collectivités veulent savoir chaque année à quelle sauce elles vont être mangées. Ce n'est pas une question de sauce : elles ne veulent tout simplement pas être mangées ! Elles sont autonomes, et le principe d'autonomie doit être respecté. Une loi de financement des collectivités territoriales serait une machine de guerre pour mettre sous tutelle les budgets des collectivités. Vous avancez un argument qui est bon, celui de l'absence de visibilité. Essayons de corriger ce problème autrement

produire un document budgétaire parfaitement limpide et clair dont nous discuterons. Mais, surtout, ne bridons pas la liberté des collectivités locales à travers un texte qui s'inspirerait du système de la loi de financement de la sécurité sociale, faite pour réduire le trou de la sécurité sociale avec des instruments très coercitifs.

Le scrutin est clos.

membres de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, des trente-six membres de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation, des trente-six membres de la délégation sénatoriale à la prospective,

58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, du chapitre 17 de l'instruction générale du bureau, les listes des candidats présentés par les groupes ont été publiées. Ces candidatures seront ratifiées si la présidence ne reçoit pas d'opposition dans le délai d'une heure.

appels d'organisations syndicales ont exprimé haut et fort, à plusieurs occasions, la revendication d'une participation accrue à la décision publique. Ces mouvements témoignent du rejet de notre modèle libéral et de la crise de confiance des citoyens à l'égard des élus. Ce constat nécessite une évolution urgente des modes de participation des citoyens pour les associer aux décisions qui les concernent et les impactent dans leur quotidien, tout particulièrement celles des collectivités territoriales. Nous ne pourrons sortir de cette crise démocratique sans replacer nos concitoyens au coeur de l'action publique. Redonner de la confiance dans l'exercice démocratique doit être notre priorité. Nous devons engager une réforme profonde de nos institutions avec une implication beaucoup plus forte au niveau local. Le référendum d'initiative locale permettrait ainsi à un nombre de citoyens résidents d'interpeller les élus locaux soit par référendum, soit par le vote de l'assemblée délibérative. Cette demande de citoyenneté active doit aujourd'hui s'inscrire dans notre Constitution, et le référendum d'initiative citoyenne doit trouver une traduction locale. Il conviendra ensuite d'en préciser les modalités dans une loi organique. Quel est l'avis de la commission ? Mon

le référendum. Or nous pensons que la démocratie représentative a toute sa valeur associée à la démocratie participative. Inverser les rôles risquerait parfois

J'espère, madame la ministre, que nous n'arriverons jamais au cinquième « D », celui de la disparition de certaines de nos collectivités territoriales, faute de moyens financiers. financiers. Il faut donner une visibilité financière aux collectivités. Il s'agit de défendre leur autonomie : toute création ou extension de compétence résultant d'une décision de l'État doit être accompagnée des ressources nécessaires. Cela va sans dire, mais les ressources attribuées doivent faire régulièrement l'objet d'un réexamen. Faisons confiance à nos élus locaux. Depuis toujours, lorsqu'ils décident, ils paient.

à M. Guy Benarroche. Depuis les années 1980, les différents gouvernements se sont efforcés d'encourager les mouvements de décentralisation. À l'heure où les collectivités manifestent leur volonté d'agir en faveur de la transition écologique et où l'action publique doit porter ses efforts en matière de justice sociale et apporter des réponses fortes à la crise démocratique que nous traversons et que j'évoquais à l'instant, il est indispensable de renforcer l'action des collectivités territoriales par une plus grande liberté fiscale et de faire de l'autonomie financière un principe constitutionnel. À mesure que nous progressons dans les mécanismes de décentralisation, nous entendons la même petite musique lancinante selon laquelle les collectivités seraient dépensières et qu'elles ne maîtriseraient pas leur budget.

en inscrivant dans la Constitution le principe d'autonomie financière, à charge ensuite au législateur d'en définir les modalités. Quel

les citoyens de l'Union européenne peuvent aujourd'hui voter aux élections locales, c'est dans le cadre d'accords de réciprocité. Votre amendement a pour

à M. Rémy Pointereau. Le 12 janvier 2016, le Sénat examinait et votait une proposition de loi constitutionnelle relative à la compensation de toute aggravation par la loi des charges et contraintes applicables aux collectivités territoriales,

visait à inscrire dans la Constitution différents principes pour inciter le législateur à accepter que lui soient fixés comme objectifs contraignants la simplification des normes et la stabilisation ou l'allégement des charges applicables aux collectivités territoriales, lesquelles sont souvent confrontées à une baisse importante de leurs ressources. Trois principes clairs

locales. Deuxième principe : la création d'un mécanisme de « gage normatif », applicable aux projets et propositions de loi comme aux amendements, obligeant à compenser toute nouvelle charge ou contrainte aux collectivités territoriales par la suppression d'une charge ou contrainte d'importance équivalente- c'est le principe du « ». Je serais Je serais même pour un « » ... Troisième principe : interdire la surtransposition de directives européennes par des textes se présentant comme des transpositions de celles-ci. Le présent amendement vise à reprendre ce dernier principe. Il n'est en effet pas rare que les projets de loi assurant la transposition des directives européennes aillent au-delà des exigences définies par le législateur européen, introduisant ainsi de manière quasi subreptice des contraintes et charges nouvelles, notamment pour les collectivités territoriales.

agacement, une irritation, à l'égard des excès de normes. Il arrive effectivement qu'au Parlement français on surenchérisse sur la norme. J'entends bien le propos.

si notre pays voulait introduire des dispositions plus fortes, plus strictes, que celles de l'Union européenne, au sein de laquelle il faudrait convaincre des pays qui n'ont pas la même vision que nous, nous ne pourrions plus le faire.

à ce que la transposition des directives européennes soit proportionnée et mesurée. Puisqu'il est question de

Les corapporteurs préconisent une refonte de la dénomination par le regroupement des collectivités situées outre-mer au sein de la catégorie « pays d'outre-mer ». Il s'agit de faire correspondre le nouveau cadre constitutionnel avec une nouvelle terminologie exempte de connotations historiques et symboliques, ce que n'est pas forcément la catégorie « collectivité d'outre-mer ». En outre, cette dénomination tient compte de l'usage de plus en plus répandu du terme « pays » s'agissant des territoires ultramarins. Elle présente aussi l'avantage d'être plus utilisée en droit comparé, ce qui doit être mis en perspective avec la demande d'une meilleure insertion régionale des collectivités.

L'article 6 répond donc bien au principe fixé par la proposition 44 des 50 propositions du Sénat pour une nouvelle génération de la décentralisation. Reste qu'il pourrait être enrichi ; tel serait le cas si la proposition de terminologie que j'ai évoquée, mais aussi d'autres dispositions Les auditions annexées au rapport précité montrent la grande hétérogénéité des aspirations, qui vont de l'autonomie et de la spécialité législative les plus avancées à l'identité législative la plus renforcée. Elles montrent aussi qu'un cadre rénové pourrait permettre de remédier à de nombreux blocages. La réunion des articles 73 et 74 de la Constitution avait pour vocation première de mettre fin à l'actuelle approche binaire pour aller vers des statuts sur mesure. Elle devait aussi conférer une dimension plus tangible aux consultations des populations, qui, en l'état, demeurent abstraites et engendrent un réflexe de crainte de l'inconnu statutaire dans certains territoires, alors même que les élus peuvent être favorables à une évolution. Comme je l'ai indiqué, cet article doit être considéré comme le signe que les auteurs de la présente proposition de loi ne souhaitaient pas écarter les outre-mer de la discussion qui nous occupe.

ce qui reste parfaitement compatible avec la mise en place d'un groupe de travail. L'article 6 de la présente proposition de loi vise à fusionner les articles 73 et 74 de la Constitution afin de créer un régime constitutionnel unique pour les outre-mer. À l'instar de bon nombre de mes collègues ultramarins, je suis très favorable à une réelle fusion des articles 73 et 74 de la Constitution et, donc, à la suppression de la logique binaire qu'ils portent.

Si l'exposé des motifs de l'article 6 tel qu'il nous est proposé entre parfaitement en résonance avec le projet statutaire guyanais- déterminer avec souplesse la part de spécialité législative et la part d'identité législative -, pour autant, sa rédaction ne me semble pas totalement satisfaisante.

Les populations ne seraient en effet consultées qu'en cas de changement de régime législatif, sur le fondement de l'article 72-4 de la Constitution, sans que l'on sache si la consultation porterait aussi sur le nouveau statut, le I du nouvel article 74 n'y faisant pas référence. Enfin, il est indispensable que le pouvoir constituant inscrive dans la Constitution des mécanismes plus simples d'extension du droit commun dans les collectivités ultramarines. Le changement du cadre statutaire ne produira tous ses effets que si la production normative, aujourd'hui beaucoup trop lourde et centralisée et victime d'un manque réel de compétences, est radicalement assouplie.

contre un mauvais texte qui nous avait été présenté ; 75 % des Guadeloupéens avaient voté contre. Depuis lors, la Martinique comme la Guyane ont choisi d'adopter le statut de collectivité unique

au Gouvernement de réviser la Constitution afin de doter la Guadeloupe d'une loi organique pour tenir compte de sa situation spécifique et singulière, et ils ont mandaté les parlementaires pour relayer cette résolution à l'occasion des séances du Parlement. Nous y sommes.

d'où l'évocation de la notion de « pays », qui peut poser, pour d'autres collectivités, des difficultés ; d'où le soutien de notre collègue à la position de sagesse

Il ne faut pas qu'un ou deux territoires prennent en otage tous les autres. Les propositions qui sont faites par Micheline Jacques, par Georges Patient, par Dominique Théophile, par tous les autres, y compris par les Polynésiens, sont telles que chacun peut choisir et même choisir de ne pas choisir ! Chacun peut rester en l'état, chacun peut évoluer ; ça peut prendre des années. C'est la raison pour laquelle la présente proposition de cohabitation des articles 73 et 74, même rédigée de manière insuffisante, est parfaitement compatible avec les amendements présentés par les uns et par les autres. Je retire cet amendement de suppression.

notamment pour donner des compétences en matière pénale aux pays d'outre-mer, parmi bien d'autres évolutions qui, selon nous,

entre les articles 73 et 74 de la Constitution, si telle est la volonté et le souhait des élus et des populations concernées. Elle atteste également qu'au sein de chacune de ces catégories, ce qu'a rappelé M. Lurel, il est tout à fait possible de retenir des modes de gouvernance, des compétences ou des instances locales propres.

que de Saint-Pierre-et-Miquelon. Quant à Wallis-et-Futuna, le Gouvernement est dans l'attente depuis de nombreuses années d'une modernisation de son statut, ne serait-ce que pour l'ériger au niveau organique. Ainsi, il ne paraît nullement nécessaire de procéder à une fusion pure et simple, comme cela est parfois proposé, pour permettre des statuts sur mesure et évolutifs. J'émets donc un avis favorable sur l'amendement n° 31. La parole

qui paraît préserver l'unicité de la République. On ne crée pas pour autant un pays fédéral, même si, avec la Nouvelle-Calédonie, on est déjà quelque part un pays archipélique.

sur la différenciation territoriale postérieures à la présente proposition de loi constitutionnelle, tout en offrant une base aux futurs travaux du groupe de travail. En prévoyant d'insérer deux articles 72-5 et 72-6 dans la Constitution, à préserver les articles 73 et 74 de la Constitution. Cette rédaction permet, sans obliger, un plus grand large champ de différenciation pour les collectivités qui le souhaitent. C'est le cas de Saint-Barthélemy. Surtout, cette rédaction vise à apporter une réponse aux aspirations expérimentées en résolvant certains blocages, en renforçant les garanties constitutionnelles portant sur la place des électeurs, le respect de leurs décisions et avis et ceux des assemblées locales. Ainsi, cet amendement tend à créer la catégorie de pays d'outre-mer et vise à organiser le maintien provisoire des articles 73 et 74, qui ne seraient abrogés à l'égard des territoires qu'avec l'entrée en vigueur du statut de pays d'outre-mer. Chacun disposerait d'un statut fixé par une loi organique dont les éléments essentiels ne pourraient être modifiés sans l'accord des électeurs, voire de l'assemblée délibérante concernée. Ce cadre permettrait une grande liberté de différenciation allant de la plus large autonomie à la plus large identité législative. L'architecture, à cette fin, serait la suivante. Premièrement, un nouvel article 72-5 comportant des éléments propres à ce statut. Il innove sur plusieurs points tels que l'impossibilité de retirer à un pays d'outre-mer, sans son accord, ses compétences particulières, ou encore en renforçant l'efficacité des procédures d'approbation de certains actes ou la démocratie locale. un nouvel article 72-6 décrivant les compétences des pays d'outre-mer en reprenant pour l'essentiel les compétences régaliennes dont l'État ne peut se dessaisir, sous réserve du cas du droit pénal spécial. Les possibilités d'association des pays d'outre-mer aux décisions les concernant en matière internationale et européenne seraient renforcées. Par ailleurs, les dispositions des articles 72, 72-3 et 72-4 sont modifiées pour tenir compte de la création des pays d'outre-mer. Conformément à l'esprit de concertation devant prévaloir à la refonte des dispositions sur l'outre-mer de la Constitution, cette proposition a vocation à être affinée. Il s'agit de prendre acte d'une direction. Attendre l'unanimité reviendrait toutefois à conférer un droit de veto à une ou à plusieurs collectivités sur les autres, ce qui est à rebours de la philosophie semblant devoir présider à cette réflexion.

comme aujourd'hui dans le, sans le sacraliser, pourraient le faire. Celles et ceux qui voudraient prendre un petit degré ou un grand degré d'autonomie, avec les responsabilités qui l'accompagnent, pourraient le faire. Ce texte est d'une grande plasticité, d'une belle audace et d'une grande beauté : je vous appelle à le voter.

le congrès des élus départementaux et régionaux pour nous permettre de débattre de toute question liée à l'évolution institutionnelle. Nous avons travaillé sur ce point pendant des années,

d'outre-mer, régies par l'article 74 de la Constitution, et aux départements et régions d'outre-mer (DROM), régis par l'article 73 de la Constitution. Les collectivités d'outre-mer deviendraient automatiquement des POM tandis que les DROM entreraient dans cette catégorie après adaptation d'un statut défini par une loi organique et après recueil du consentement des électeurs intéressés.

À titre d'exemple, les amendements visent à prévoir que le statut des POM leur permet d'exercer un pouvoir normatif autonome dans le domaine de la loi ou du décret, ou de subordonner l'adoption de dispositions particulières relatives à ces collectivités à l'accord de leurs institutions. Cela revient à constitutionnaliser un domaine réservé que le législateur ne pourrait plus modifier sans leur accord. Ensuite, ils visent qu'un pays d'outre-mer peut être membre d'une organisation internationale, disposer d'une représentation auprès d'États ou d'organisations internationales, négocier des accords

d'outre-mer. Je ne suis pas sûre que tout le monde soit complètement d'accord. Un département comme Mayotte, très attaché à son statut, qui ne souhaite pas

Si, en tout état de cause, il fallait avancer vers une évolution systémique, la plus importante depuis 2003, il convient de mettre en place une large concertation avec les élus et l'ensemble des territoires concernés. concernés. Je rejoins donc la proposition du sénateur Mathieu Darnaud : si votre intuition est bonne, il faut la confronter

J'ai également entendu la position du corapporteur, mais je suis convaincue que la démarche consistant à vouloir inclure les outre-mer dans cette proposition de loi constitutionnelle est conforme aux prérogatives du législateur et fait écho à la réalité du territoire de la République dans son ensemble. Je suis attachée à ce que des dispositions outre-mer figurent dans ce texte. Cela me semble d'autant plus important que la création des articles 72-5 et 72-6 tend à maintenir en l'état les articles 73 et 74 de la Constitution. Il faut donc y voir une ouverture du champ des possibles pour les collectivités qui le souhaitent, sans remise en cause de l'existant pour celles qui ne le souhaitent pas. En cela, la dénomination de pays d'outre-mer est un point qui pourra faire l'objet de discussions, d'autant qu'elle n'est pas incompatible avec les actuelles incompatible avec les actuelles dénominations de départements et de régions. À cet égard, la Polynésie française, tout en étant une collectivité d'outre-mer, est un pays d'outre-mer au sein de la République. Il s'agit donc de prendre acte des aspirations qui se sont exprimées dans le respect des volontés de celles des collectivités qui sont favorables au et de prendre date. Un travail d'élaboration d'un texte définitif pourra se poursuivre. Pour ces raisons, je maintiens l'amendement n° 9 rectifié, et j'espère que mes collègues le voteront. La parole est à M. Philippe Bas, pour explication de vote. explication de vote. Je dois vous rendre compte du travail accompli au sein du groupe de travail mis en place par le président Larcher au début de cette année, travail auquel a été associé très étroitement M. Michel Magras, alors président de la délégation sénatoriale

très nombreux contacts pris par Michel Magras que les dispositions inscrites dans cette proposition de loi constitutionnelle ont été arrêtées par notre groupe de travail. Ces dispositions avaient pour objet d'assouplir les règles constitutionnelles applicables à nos collectivités d'outre-mer en effaçant une distinction dont nous avons considéré collectivement qu'elle n'avait plus de raison d'être

des situations. J'ai donc examiné avec un peu de perplexité les amendements dont nous discutons actuellement. Je reconnais leur mérite, ce sont des amendements qui ont été travaillés

n'a pu être conduite de manière approfondie. Si nous voulons faire du bon travail, mieux vaut ne pas adopter ces amendements, non que nous les rejetterions sur le fond, ce qui n'est pas le cas, mais parce que nous avons besoin d'un travail complémentaire et d'une concertation plus forte. Il y a ici trop

Saint-Martin ne souhaite pas, contrairement à d'autres collectivités ultramarines, se voir transférer l'ensemble des compétences à l'exception du pouvoir régalien de l'État. Pour rappel, notre statut de collectivité d'outre-mer (COM) dotée de l'autonomie est relativement récent puisqu'il a Notre priorité dans le contexte économique, social et sanitaire difficile actuel est d'optimiser les outils juridiques, administratifs et institutionnels permettant de consolider notre reconstruction post-Irma, d'engager notre relance de l'après-covid-19 et ainsi de réussir le développement durable et solidaire de Saint-Martin. Les lignes de partage entre l'État et la COM fixées par la Constitution et notre loi organique de 2007 sont plutôt claires et nous conviennent globalement, ce qui n'exclut pas à l'avenir des ajustements législatifs permettant d'améliorer les dispositions de notre statut. de notre statut. Pour nous, le point de vigilance n'est pas le débat statutaire, mais est la juste pratique institutionnelle. Pour autant, des pistes d'amélioration existent. Il est en effet possible et souhaitable d'améliorer le statut constitutionnel des outre-mer en remédiant notamment aux difficultés et aux blocages constatés dans la mise en oeuvre des réformes constitutionnelles de 2003 et de 2008. Les amendements présentés par Micheline Jacques et par mes autres collègues constituent une bonne base de travail pour le futur. Il est donc nécessaire que l'article 6 soit retiré.

tout en opérant une mise à jour du préambule de la Constitution afin qu'il corresponde à la situation actuelle des outre-mer, qui a évolué depuis 1958. La création de la catégorie des pays d'outre-mer étant conçue pour permettre une évolution différenciée, il convient de l'assortir d'une affirmation au niveau des dispositions les plus solennelles et symboliques, précisant que cette réforme n'implique en rien un risque de distanciation des liens de citoyenneté au sein du peuple français. Il s'agit d'affirmer que le statut des pays d'outre-mer, qui tient compte de leur intérêt propre au sein de la République, comporte des éléments constitutifs qui ne pourraient être modifiés sans leur accord. Il vous est ainsi proposé de constitutionnaliser l'obligation de recueillir le consentement des populations pour toute éventuelle séparation d'avec la République. Une telle hypothèse exigerait une révision de la Constitution. Ainsi, une éventuelle séparation ne pourrait pas seulement résulter d'une loi organique. Il s'agit, de plus, de consacrer pleinement le droit à la libre détermination, mais en le déconnectant des traités internationaux prévus à l'article 53, alinéa 3, de la Constitution.

que le caractère historique que vous appelez de vos voeux ne se retrouve pas au terme du processus et de la réflexion que nous mènerons en commun. Quel

de recourir aux ordonnances, afin d'y appliquer ou d'y adapter les dispositions législatives après avis des assemblées délibérantes. Ces ordonnances doivent faire l'objet, à peine de caducité, d'une ratification expresse par le Parlement dans un délai de dix-huit mois suivant leur publication. Techniquement, ce dispositif est indépendant des propositions présentées par ailleurs s'agissant de la substitution progressive des « pays d'outre-mer » aux actuels DROM et COM. Il peut donc être adopté indépendamment de cette évolution globale du cadre constitutionnel des outre-mer, Nouvelle-Calédonie. Il s'inscrit, pour autant, dans la même démarche, qui vise à accélérer autant que possible l'actualisation du droit des outre-mer. À cette fin, l'objet des ordonnances est expressément étendu à la codification et à l'actualisation des dispositions en vigueur, en vue d'assurer le respect du principe de la hiérarchie des normes et de renforcer leur intelligibilité. par ailleurs, d'accélérer autant que possible la ratification de ces ordonnances appelées à être plus nombreuses, eu égard à la multiplication des statuts particuliers, mais aussi de permettre une plus grande réactivité du Parlement en matière d'actualisation du droit des outre-mer, et à cet effet d'adoption, d'approbation ou de ratification des textes pour lesquels les nouvelles lois organiques prévoiraient un contrôle parlementaire. Il est proposé de constitutionnaliser la possibilité de recourir à des procédures d'examen simplifié, telle que la procédure de législation en commission ; les règlements des assemblées parlementaires détermineraient les conditions dans lesquelles il pourrait y être recouru. Cette procédure serait prévue pour l'adoption des projets et propositions de loi ayant pour principal objet la modification des dispositions législatives applicables outre-mer, ou la ratification d'ordonnances ou de décrets y afférents. Ce dispositif met également en oeuvre l'une des préconisations du rapport de la délégation sénatoriale aux outre-mer sur la différenciation territoriale.

du législateur les dispositions en vigueur dans les collectivités ultramarines. Une telle possibilité, en effet, aurait pour conséquence de dessaisir le législateur de larges pans du droit. Le sous-amendement tend également à supprimer la disposition selon laquelle le règlement des assemblées parlementaires détermine les conditions dans lesquelles il est recouru à des procédures simplifiées pour l'adoption des textes ayant pour objet les collectivités ultramarines ou la ratification d'ordonnances y afférentes. Le recours à de telles procédures est déjà possible et doit demeurer facultatif en fonction des enjeux des différents textes. Quel est

que la différence de traitement se justifie historiquement, puisque les collectivités d'outre-mer sont régies par le principe de spécialité législative, et elle présente un enjeu constant d'extension ou d'adaptation de mesures législatives nationales. cette habilitation permanente permet une souplesse. Étendre cette habilitation aux DROM peut se comprendre : ce serait un gage de rapidité et d'efficacité. Toutefois, il semble difficile d'y être favorable- j'en suis désolée, monsieur Lurel -en l'absence d'une concertation avec les DROM. Ceux-ci pourraient en effet avoir le sentiment que nous allons adapter leur droit par ordonnances, sans accord de leur part.

d'adaptation, prévu à l'article 73 de la Constitution. Ils peuvent demander au Gouvernement ou au Parlement de les habiliter à déroger à la loi ou au règlement au titre soit de leurs compétences, soit de celles de l'État. À cet égard, le projet de loi constitutionnelle porté par le Gouvernement prévoyait de simplifier drastiquement

puisse se dérouler sur la durée d'une mandature. Pour le reste, nous dépendons du bon vouloir de l'administration lorsqu'il s'agit de décrets. Quant au Parlement, quelquefois il ne répond pas. Il faut améliorer les choses et continuer à se battre.

certaines avancées : la clause générale de compétence des communes, l'assouplissement des modalités d'expérimentation, la différenciation des compétences, la différenciation normative et l'autonomie financière.

et il votera de grand coeur cette proposition de loi constitutionnelle. J'en suis particulièrement ému. Une nouvelle étape s'ouvre. Je souhaite vivement que ce texte soit adopté à une très large majorité et qu'il puisse être rapidement débattu à l'Assemblée nationale. Il n'y a pas

En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit. Il va y être procédé dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert.

en termes d'aménagement du territoire. Actuellement, les études d'impact ne mesurent que les conséquences économiques, financières, sociales et environnementales des projets proposés. Trop de réformes, notamment dans les domaines de la santé, du numérique et de la réorganisation territoriale, ont été menées

à évaluer l'ensemble des incidences techniques et financières des mesures proposées, selon leur nature et le mode de financement dans les domaines de compétences, sur l'emploi et sur les politiques mises en oeuvre. Par ailleurs, la rubrique de l'étude d'impact dédiée à l'analyse des impacts environnementaux doit d'ores et déjà faire apparaître, si le sujet le justifie, outre le coût des mesures envisagées pour le climat et pour la biodiversité, les incidences du projet de loi sur les territoires, la mobilité des personnes ou des marchandises, la consommation d'énergie et le niveau de production des entreprises. Beaucoup d'éléments

pour objet de rétablir le caractère limité de la durée des expérimentations, laquelle est actuellement fixée à cinq ans par le premier alinéa de l'article L.O. 1113-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). La limitation de cette durée est inhérente au principe même d'expérimentation. En effet, l'expérimentation doit conserver une durée limitée pour qu'il puisse être établi, à son issue, s'il est nécessaire de proroger l'expérimentation sur tout ou partie du territoire, ou s'il est préférable de l'abandonner. En outre, l'article L.O. 1113-6 du CGCT permet déjà au législateur ou au pouvoir réglementaire qui autorise une expérimentation de la prolonger pour une durée pouvant aller jusqu'à trois ans,

Or, dans un objectif de simplification, il ne semble pas utile que ce rapport intègre un bilan annuel de l'ensemble des expérimentations, dès lors que le premier alinéa de l'article que j'ai que le Gouvernement transmet au Parlement, pour chaque expérimentation réalisée et avant l'expiration de sa durée, un rapport d'évaluation

Au nom de la simplification, vous nous proposez de supprimer l'exercice, alors qu'il nous semble extrêmement important, si nous nous engagions dans une loi de décentralisation incluant de la différenciation,